reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.-

est apparue parallèlement au développement des techniques de procréation médicalement assistée. Le projet parental, c'est le fait de souhaiter un enfant. Si un tel souhait suffit à légitimer l'accès à la PMA, il s'agit alors d'un droit à l'enfant, même s'il faut noter que l'expression « projet parental » évacue le terme « enfant » au profit de celui Par son aspect volontairement flou, ce concept ouvre un champ des possibles quasiment infini : l'autoconservation de gamètes sans motif médical,

Il s'agit d'un amendement de coordination par anticipation avec un amendement que nous avons déposé à l'article 3, et qui tend à préserver l'anonymat du donneur dans le cadre de la procréation médicalement assistée. objet est clair : souligner les conséquences problématiques de la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes. Je précise qu'il n'est question que du nom du donneur, pas d'informations génétiques utiles aux donneurs comme aux enfants nés du don.

Or cette faculté, si elle est confortable pour le donneur, est plus discutable du point de vue des enfants. Elle les placerait dans une situation d'inégalité selon le choix du donneur. Surtout, l'utilité de cette disposition n'est pas convaincante. On comprend aujourd'hui la nécessité que ressentent les enfants issus de dons de gamètes de connaître leurs origines. C'est une quête tout à fait compréhensible qu'ils partagent avec la plupart de nos concitoyens, si l'on en croit l'engouement pour la généalogie. contribue à la construction de l'identité narrative, comme l'appelait Bourdieu, de tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie. S'agissant du don de gamètes, nous craignons que la levée de l'anonymat ne charge de sens familial un acte qui s'en éloigne absolument. nous considérons que l'essentiel de la filiation se manifeste après la naissance, dans l'éducation, les soins et l'affection apportés, ainsi que dans les valeurs transmises. Il est possible que plus le mystère de la conception soit grand, plus la quête des origines soit impérieuse.

Pour être clair, il s'agit de permettre à des enfants, à l'âge de 18 ans, d'accéder à leurs origines, à des données soit anonymisées, soit non anonymisées.

Mme Michelle Gréaume. Il semblerait que le fil rouge des réformes judiciaires des années 2000 soit la déjudiciarisation, laquelle est surtout conçue et recherchée pour les économies de tout ordre qu'elle permet.

Un certain nombre d'articles, notamment ceux qui sont relatifs à la PMA, confient aux notaires des pouvoirs jusqu'ici du ressort des juges et de l'officier d'état civil. Il s'agit d'un pas de plus vers la déjudiciarisation de la famille qui ne cesse de s'accentuer depuis les années 1960. en France, la tendance est à la déjudiciarisation de tout ce qui ne suscite pas de conflits : divorce par consentement mutuel, PMA de couples lesbiens, etc. La prochaine étape concernera peut-être l'adoption.

En outre, les nouvelles compétences accordées aux notaires semblent assez mal reçues par la profession elle-même, qui considère notamment que les questions de filiation sont extrêmement importantes,

pour le notaire, le reste étant réservé à l'enregistrement et à la conservation de l'acte. Il s'agira vraiment d'un service social, a déclaré maître Bertrand Savouré lors de la réunion que j'ai précédemment mentionnée. Tous ces éléments nous conduisent à penser qu'il est absolument nécessaire que cet acte soit du ressort du juge.

Le nouvel article L. 2141-6 du code de la santé publique prévoit qu'un couple ou une femme non mariée souhaitant accueillir un embryon doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, dans les conditions prévues par le livre I du code civil.

madame la ministre

Je rappelle que ces couples donneurs d'embryons font déjà l'objet d'une sélection médicale rigoureuse. Ainsi, à l'échelon réglementaire, les critères médicaux d'acceptabilité ont été définis et des tests de sécurité sanitaire sont réalisés, ainsi qu'une étude de risques génétiques des deux membres du couple.

il s'agit non seulement d'étendre la PMA à toutes les femmes, mais aussi, par exemple, d'autoriser l'autoconservation des gamètes. Ces nouvelles dispositions impliquent de déployer des moyens, sans parler de la nécessité de faire appel aux dons, bien sûr,

L'exploitation des gamètes par des établissements privés à but lucratif livre la procréation au marché. Cela entre en totale contradiction avec le principe bioéthique français de non-marchandisation du corps, auquel nos concitoyens sont très attachés. Il semble important de répondre aux besoins dans le domaine du don de gamètes, mais il faut faire en sorte que les principes éthiques ayant toujours fondé nos lois de bioéthique soient préservés. J'ajoute qu'étendre à des centres privés l'habilitation à l'autoconservation constituerait un facteur majeur d'inégalités. Seules les personnes aisées y auront accès, ce qui améliorera leur carrière par report des projets parentaux et, donc, augmentera encore davantage les inégalités sociales dans notre pays.

La pénurie annoncée de gamètes laisse augurer une importation de sperme depuis l'étranger ou une rémunération des donneurs, mesure suggérée par certains gynécologues. exploités par des établissements privés à but lucratif démontre que des intérêts commerciaux importants sont en jeu et que la procréation peut être insidieusement livrée au marché, en contradiction avec le principe bioéthique français de non-marchandisation du corps.

l'article 1, tel qu'il découle des travaux de la commission spéciale, permet d'ouvrir l'activité de conservation d'embryons aux centres privés à but lucratif. Loin de moi l'idée de remettre en cause la compétence de ces établissements, qui sont soumis aux mêmes conditions d'éthique médicale, d'autorisation et de contrôle que les centres publics ou privés à but non lucratif. J'entends également l'argument de la commission spéciale, selon laquelle cette mesure permettrait notamment de réduire les délais importants dans l'accès à l'assistance médicale à la procréation et d'assurer une certaine égalité territoriale. Pour autant, comme l'a rappelé Mme la ministre lors des débats à l'Assemblée nationale, seulement 19 centres, publics ou privés à but non lucratif, sont autorisés à exercer et seulement 19 transferts d'embryons de parents donneurs vers des parents candidats pour les accueillir ont été comptabilisés en un an.

Cette dernière, qui ne présente pas de difficultés techniques particulières, ne s'est jamais développée à hauteur des espérances, en raison de la difficulté de la démarche pour les couples concernés, notamment sur le plan psychologique, qu'ils soient en situation de donner ou en situation d'accueillir un embryon.

de me risquer à faire un peu de pédagogie schématique ... En matière d'AMP, trois types de centres interviennent : les centres publics, les centres privés à but non lucratif et les centres privés à but lucratif. Il y a, schématiquement, trois sortes d'activités

Les trois types de centres peuvent tout faire, à l'exception de l'accueil d'embryons et du don de gamètes, dont sont exclus les centres privés à but lucratif, pour des motifs que Mme la ministre des solidarités

C'est pourquoi je suivrai la commission

des embryons dont le plus grand nombre est destiné à la destruction par arrêt de conservation, et dont d'autres pourront être utilisés, avec l'accord

c'est l'existence d'une préoccupation publique de sécurité sur la manière dont ces embryons vont être conservés,

aujourd'hui du ressort du secteur public et du privé non lucratif, pour des raisons fondamentales de bioéthique, en particulier la non-marchandisation du corps humain et de tous les produits du corps humain,

couvertes par les centres publics. À ce stade, je souhaiterais que le débat se cantonne aux embryons, puisque nous aurons l'occasion de reparler du don et de la congélation de gamètes. cette ouverture au secteur privé, non parce que nous stigmatisons telle ou telle activité, mais parce que c'est un principe fondamental de la bioéthique que de ne pas confier des morceaux du corps humain au secteur privé.

pour concevoir l'embryon qui sera implanté dans l'utérus de la femme, dans l'intérêt de l'enfant. Cette pratique de l'AMP avec don de gamètes, très minoritaire,

L'interdiction du double don de gamètes devrait être maintenue, le double don n'étant d'aucune utilité dès lors que la possibilité d'accueillir un embryon est autorisée. Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA,

que l'équipe médicale qui entoure ces couples infertiles comprend un certain nombre de professionnels de santé capables d'évaluer le couple dans son entièreté, si je puis dire, en termes de capacités d'accueil de l'enfant.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement tend à supprimer la mention adoptée en commission spéciale et visant à rappeler « les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ». L'assistance médicale à la procréation est un parcours lourd, difficile et réfléchi. Nous considérons, bien qu'attachés à ce qu'une information complète soit donnée au demandeur souhaitant procéder à un parcours d'AMP, que cet ajout introduit un jugement de valeur face à la démarche souhaitée. Par ailleurs, il serait difficilement envisageable pour l'équipe médicale d'établir une relation de confiance si l'un des premiers éléments imposés est de rappeler que leur démarche n'est pas la bonne. Il n'est pas ici question de dissuader le demandeur et c'est, en quelque sorte, ce qui est induit par cette précision. Quel est l'avis de la commission spéciale

Nous considérons, en premier lieu, que l'introduction de la mention de « l'évaluation psychologique et sociale » pose question au moment où nous nous apprêtons à voter le droit pour toutes à l'AMP. Certes, l'évaluation psychologique concernerait tous les couples, hétérosexuels ou lesbiens, ainsi que les femmes seules. Nous savons également qu'elle existe pour les couples souhaitant adopter un enfant. Néanmoins, nous estimons que cela ne doit pas guider l'élaboration du dispositif d'AMP. En effet, un couple ou une femme non mariée souhaitant recourir à l'AMP n'ont pas à être différenciés d'un couple hétérosexuel décidant de faire un enfant sans avoir recours à cette technique. Dans ces trois cas, il s'agit d'un même projet parental. Aussi, nous ne saisissons pas les raisons pour lesquelles, dans le cas où le projet s'inscrit dans le cadre d'une AMP, le couple ou la femme devrait subir une évaluation autre que médicale. Cela serait stigmatisant pour ces personnes et dommageable dans la procédure de l'AMP.

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que l'introduction de ce type d'évaluation a un lien avec le projet parental d'un couple de femmes ou d'une femme seule, même indirect. Faut-il encore rappeler, à ce stade du débat, que les enfants issus d'une PMA, notamment ceux qui ont pour parents deux mères, ne sont pas moins épanouis ou plus épanouis que les autres. Je renvoie à toutes les études qui ont été réalisées sur ce sujet. En second lieu, il nous semble très important, surtout au vu de nos discussions, que la loi garantisse expressément au sein du dispositif le principe de non-discrimination, en énonçant les motifs qui pourraient conduire une équipe médicale à refuser l'AMP à un couple ou à une femme seule. Pour finir, nous regrettons que ce projet de loi, alors même qu'il constitue une avancée sociale importante, avec l'ouverture de la PMA pour toutes, contienne encore des dispositions discriminatoires qui traduisent une suspicion à l'égard des couples lesbiens et des femmes non

elle pourrait donner le sentiment que l'accès à l'AMP est conditionné à une procédure d'agrément et susciter des inquiétudes, à juste titre. Prenons l'exemple de la polémique récente concernant l'adoption des couples homoparentaux. La présence d'un psychiatre ou d'un psychologue spécialisé au sein de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire est suffisante pour procéder à l'évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ayant un projet parental. Cette notion de projet parental s'entend, selon le Conseil d'État, comme incluant tant le projet familial des parents que l'ensemble des conditions propres à garantir l'intérêt de l'enfant. De ce fait, il s'agit bien ici de s'assurer que le couple ou la femme non mariée pourra subvenir aux besoins de l'enfant.

Dans le cadre d'une procédure d'adoption, une enquête sociale et psychologique est imposée aux postulants. Cette enquête vise à déterminer les garanties que la famille peut offrir à l'enfant : capacités morales, éducatives, affectives, familiales et psychologiques.

la présence d'un psychologue dans l'équipe pluridisciplinaire qui reçoit les couples demandeurs à l'AMP. Le projet de loi mentionnait également cette évaluation psychologique. L'Assemblée nationale l'a supprimée, tout en maintenant la présence d'un psychologue. Nous tirons les conséquences de la présence du psychologue dans cette équipe en indiquant qu'il sera procédé à une évaluation psychologique. Voilà quelle est la logique.

la possibilité de procéder à une évaluation sociale « en tant que de besoin ». Autrement, rien ne justifie la présence de ce travailleur social. Nous l'avons introduite « en tant que de besoin », parce qu'elle ne doit pas être réalisée systématiquement. Ce sont les équipes qui estiment si, oui ou non, et encore une fois, quel que soit le public concerné, il est nécessaire de procéder à cette évaluation sociale, sans que cela soit discriminant. Voilà pourquoi la commission a ainsi rédigé son texte. Elle émet un avis défavorable sur les dispositions qui y contreviennent. Quant au rétablissement d'une référence que nous avons supprimée après son adoption à l'Assemblée nationale, selon laquelle cette évaluation du couple ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son

à l'assistance médicale à la procréation. En effet, c'est le rôle de l'équipe clinicobiologique qui peut, si elle l'estime nécessaire, faire appel à un assistant social. Cela est très clairement précisé dans le projet de loi, à l'alinéa 35, soit besoin de le répéter. Introduire une évaluation sociale alors que nous ouvrons l'AMP à de nouveaux publics laisse entendre aux intéressées

ne pas mettre en oeuvre la procédure d'assistance médicale à la procréation, notamment lorsque, « après concertation au sein de l'équipe [ ...], il estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l'intérêt de l'enfant à naître vous le voyez bien : il n'y a pas de droit d'accès illimité et absolu à l'assistance médicale à la procréation, quels que soient d'ailleurs les demandeurs. Alors que

Mme la ministre.

Dans l'intérêt de l'enfant, le Gouvernement a entendu faciliter, par ce projet de loi, l'accès aux origines.

d'un don constitue un préalable logique à la recherche des origines que lui seul décidera ensuite, à sa majorité, d'entreprendre ou non.

de son mode de conception. C'est pourquoi nous proposons que les parents soient sensibilisés à cette question, dans le cadre de leur parcours d'AMP. Il s'agirait d'inscrire dans le dossier guide remis par le médecin aux couples ou aux femmes seules des éléments quant à la nécessité d'anticiper et, ce faisant, de créer des conditions permettant de faire savoir à l'enfant, avant sa majorité, qu'il est issu d'un don. Cette mention écrite serait renforcée par une information orale.

Le dernier alinéa du nouvel article L. 2141-10 du code de la santé publique dispose que le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. Cet amendement tend à ouvrir la possibilité pour le couple et la femme non mariée de donner, dans les mêmes conditions, leur consentement à un avocat.

a souhaité réserver aux seuls couples de sexes différents le remboursement par la sécurité sociale de l'AMP avec tiers donneur : elle a clairement voulu non pas exclure les couples lesbiens et les femmes seules

l'amendement n° 262 rectifié. Dans sa rédaction initiale, l'article 1 garantissait l'égal accès aux techniques de procréation médicalement assistée pour l'ensemble des femmes, que leur impossibilité d'avoir un enfant soit liée à une infertilité ou à leur situation personnelle. Par la prise en charge intégrale de l'AMP par l'assurance maladie, ce texte rendait donc réel l'accès à un droit étendu. il est regrettable que la commission spéciale ait réduit le champ de la prise en charge aux couples hétérosexuels et selon un critère pathologique. Premièrement, la mise en oeuvre de l'AMP pour les couples hétérosexuels ne s'inscrit pas toujours, en pratique, dans un contexte pathologique. Deuxièmement, comme le rappelle le Conseil d'État, « l'équité

dans les faits, entre ressources économiques et concrétisation du projet parental des couples de femmes et des femmes seules. Troisièmement et enfin, alors que la question des coûts ne saurait constituer le critère ultime

reconnaître dans la loi la légitimité d'un projet parental tout en le privant, en pratique, des conditions de sa réalisation nous paraît peu soutenable. C'est pourquoi nous proposons par cet amendement de réintroduire la prise en charge de l'AMP pour l'ensemble des couples hétérosexuels ainsi que pour les couples de femmes et les femmes seules.

accompagné et à l'issue d'une évaluation médicale. Le cadre sera exactement le même pour les couples de femmes et les femmes non mariées. La commission spéciale a souhaité réserver la prise en charge de l'assistance médicale à la procréation par l'assurance maladie aux seuls couples hétérosexuels infertiles.

Une des priorités des politiques publiques est de chercher à limiter les inégalités sociales liées aux revenus : le Gouvernement ne pourrait se résoudre à ouvrir un droit qui serait réservé aux femmes les plus aisées. En tout état de cause, le Conseil d'État a tranché la question par son étude de juin 2018 : « Il paraît exclu, pour des raisons juridiques, d'établir un régime différent de prise en charge au regard de la seule orientation sexuelle. » Voilà pourquoi nous entendons revenir au texte initial : nous ne souhaitons pas aboutir à un droit formel, qui ne serait pas un droit réel.

peut-être faire du droit ... Ainsi, pour savoir les actes qui doivent être remboursés par la sécurité sociale, nous nous référons au code de la sécurité sociale et aux conditions de prise en charge de ces actes,

L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple formé d'un homme et d'une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. » Il me semble que nous nous trouvons là dans les conditions de remboursement fixées par le code de la sécurité sociale.

Conseil d'État. C'est important : il est vrai que le Conseil d'État a indiqué qu'il paraissait exclu, pour des raisons juridiques, d'établir un régime différent de prise en charge au regard de la seule orientation sexuelle. point, je vous rejoins. Toutefois, il a également précisé : « Le seul critère pertinent serait la visée thérapeutique, à l'instar de ce qui existe pour distinguer la chirurgie esthétique de la chirurgie réparatrice. » C'est toute la différence que nous souhaitons mettre en place.

et ne sont pas justifiés par une situation médicalement constatée. Il est évident que, si l'on n'a pas trouvé médicalement la cause de l'infertilité, cette été constatée. Si les couples se soumettent au traitement de l'infertilité, dont chacun a pu rappeler qu'il s'agissait d'un traitement particulièrement pénible dans un certain nombre de cas, c'est bien qu'ils ne parviennent pas à avoir d'enfant. Nous sommes

en aucun cas d'une indication médicale. Vous pouvez décider, parce que vous êtes le Gouvernement, parce que vous avez une majorité à l'Assemblée nationale, de mettre en place un financement solidaire ; personnellement, je m'y opposerai,

la mission de la sécurité sociale est, à mon sens, d'apporter ces soins et de les prendre en charge. J'entends la cohérence du raisonnement de ceux qui s'opposent à cette extension de la PMA et donc à son remboursement, mais vous ne pouvez pas nier que la conséquence très directe de ce choix, c'est que les personnes concernées vont se répartir en deux catégories

aux argumentations qui ont été présentées par mes collègues, en particulier Laurence Rossignol et Bernard Jomier. Citons quelques chiffres

à la première que, pour des raisons physiologiques, il fallait qu'ils s'y prennent d'une certaine manière pour obtenir le succès. Ils ont eu cinq enfants ... Un premier exemple de procréation médicalement assistée

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Mes chers collègues, nous avons examiné 56 amendements au cours de la journée ; il en reste 207 à examiner sur ce texte.